madame la présidente. La séance est reprise. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mercredi 21 juillet, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, en lieu et place de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique et sur le projet de loi organique modifiant la loi du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Acte est donné de cette demande.

également sur les risques psychosociaux liés à l'activité professionnelle, pour prendre en compte tant la santé physique que la santé mentale des travailleurs. Depuis plusieurs années, les études montrent que ces risques et leurs incidences sur la santé des travailleurs peuvent concerner toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Avec la pandémie, l'importance et la visibilité des risques psychosociaux se sont accrues : en mai 2020, en mai 2020, ils sont devenus la deuxième cause d'arrêt de travail, soit 12 % des arrêts, après la covid-19 et devant les troupes musculo-squelettiques. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose donc, par cet amendement, d'inclure l'analyse des facteurs de risques psychosociaux, notamment liés aux organisations du travail, auxquels sont exposés les salariés dans l'évaluation des risques dont l'employeur a la responsabilité. Quel est l'avis de la

Poncet Monge, pour présenter l'amendement n° 43. La législation relative à la reconnaissance de la souffrance au travail est au point mort depuis de nombreuses années, malgré l'explosion du nombre de maladies professionnelles nouvelles. À l'image de la recrudescence de phénomènes de burn-out, de bore-out, ou encore de la résurgence de risques psychosociaux depuis le confinement soudain des Français, le législateur aurait eu matière à agir pour mieux protéger celles et ceux qui travaillent. Nous regrettons que cette proposition de loi, pourtant le premier véhicule législatif sur la santé au travail depuis des années, ne parle précisément pas de la souffrance au travail et de ses causes profondes, notamment en s'attaquant à l'intensification de la charge de travail et à la grande pénibilité de certaines professions. Cet amendement vise à permettre aux services de prévention et de santé au travail, ou SPST, des entreprises de prendre en compte la charge de travail des salariés et la pénibilité de leur poste

les individus. Dans le monde du travail, plusieurs facteurs de risque favorisent la survenance de violences sexistes et sexuelles : conditions de travail précaires, qui se traduisent notamment par des contrats à durée déterminée

Mme Laurence Cohen. Le document unique prévu à cet article pour recenser les risques professionnels dans l'entreprise est un document important, à condition que le comité social et économique, le CSE, contribue systématiquement et préalablement à son élaboration. Depuis la fusion, en 2017, des délégués du personnel, des comités d'entreprise et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, en une instance unique, les prérogatives des représentants des salariés ont été profondément réduites. On leur demande toujours plus avec de moins en moins de moyens

est l'avis de la commission ? La loi est déjà impérative dans sa formulation. L'adverbe « obligatoirement » ne se justifie donc pas. Par ailleurs, l'évaluation des risques professionnels est un processus continu au sein de l'entreprise : le CSE doit ainsi y contribuer, en application de l'article L. 2312-9 du code du travail, en amont de la finalisation du DUERP par l'employeur. Il sera également systématiquement consulté sur le document unique et ses mises à jour et pourra formuler

il n'est pas opportun de formaliser à l'excès le processus de consultation du CSE par l'employeur en imposant la définition d'un calendrier négocié : sachons faire confiance à l'esprit de dialogue au sein des entreprises sur des sujets qui doivent rassembler la communauté de travail.

tiendra compte de l'évaluation passée. Attention de ne pas confondre le DUERP et les actions qui doivent en découler : ces dernières seront déclinées, soit dans le programme annuel de prévention, qui comprendra d'ailleurs des indicateurs de résultat pour tirer le bilan de leur mise en oeuvre,

individuelle des risques chimiques auxquels sont exposés les salariés, notamment par l'établissement d'une liste actualisée des travailleurs concernés et en répertoriant la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents chimiques. À la suite des ordonnances Travail de 2017, l'employeur n'est plus tenu à ces deux obligations, alors que le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux ou cancérigènes concerne 12 % des salariés français. raison pour laquelle le présent amendement vise à rétablir l'obligation de l'employeur de tenir à jour une liste des salariés exposés à des agents chimiques dangereux, ainsi que l'obligation d'établir une fiche

continuent d'être déclarés systématiquement par l'employeur au service de santé au travail. Ces travailleurs font également l'objet d'un suivi individuel renforcé, avec un examen médical à l'embauche, renouvelé au moins tous les quatre ans, et avec, dans l'intervalle, une visite intermédiaire effectuée par un professionnel de santé, au plus tard deux ans après la dernière visite du médecin du travail. Enfin, la commission a renforcé, à l'article 12, les données d'exposition qui devront être consignées dans le dossier médical de santé au travail, le DMST, par les professionnels de santé des SPST.

des mesures de prévention. Il doit veiller personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou réglementaires. L'amendement

qui regroupe des salariés des services de prévention, d'un risque de transfert ou, du moins, d'une dilution de la responsabilité personnelle de l'employeur, qui serait transférée vers le comité social et économique, le salarié référent et, surtout, le service de prévention et de santé au travail. Dans la droite ligne d'une jurisprudence ancienne et constante qui précise qu'il appartient à l'employeur de veiller personnellement à la stricte application, par ses subordonnés, des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel, nous proposons par cet amendement d'inscrire dans la loi que l'employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l'évaluation des risques. La proposition de loi n'acte aucun droit nouveau pour les salariés. L'employeur garde seul le pouvoir d'organisation ; il doit donc garder seul la responsabilité.

les salariés référents en santé et sécurité au travail et le SPST sont mobilisés pour apporter leur aide à l'employeur dans l'évaluation des risques professionnels et non pour se substituer à lui dans cette démarche. Il en va de même pour les méthodes et outils proposés par les organismes et instances de branche afin d'accompagner l'employeur. Madame Poncet Monge, si vous pouvez considérer qu'il n'y a aucun droit nouveau pour les salariés, je puis vous garantir qu'il n'y a aucune minoration des obligations de l'employeur,

ans. Les outils numériques nous permettent désormais de renforcer la conservation de ce document. Pour autant, il est important que les moyens d'assumer cette conservation digitalisée restent de la responsabilité de l'employeur.

prévues par décret. Par ces modifications, la conservation et l'archivage de ce document clé seront assurés de manière efficace pour tous les employeurs, au profit des salariés. Quel

tendent à revenir sur le principe du dépôt dématérialisé du DUERP sur une plateforme numérique administrée par les organisations patronales. Or sa conservation sous un format digitalisé par l'employeur ne permet pas d'envisager celle-ci sur une durée suffisamment longue pour l'ensemble des entreprises, pour

La transmission du DUERP au SPST ne doit pas être facultative, car ce document est, selon nous, capital pour permettre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire de disposer d'informations complémentaires à la fiche d'entreprise, et retracer, au fil du temps, les risques auxquels les salariés ont pu être exposés. Enfin, la responsabilité de l'élaboration du DUERP pèse uniquement sur l'employeur. Par conséquent, il n'apparaît pas opportun de transférer aux SPST l'obligation de sa conservation et de sa mise à disposition, dès lors que seul l'employeur reste maître de sa transmission. La

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à intégrer l'avis du CSE aux éléments que l'employeur se doit de transcrire dans le DUERP. L'article 2 prévoit de renforcer l'implication du CSE,

dans l'élaboration du DUERP. Il précise que ces acteurs contribuent à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise, et que le comité social et économique est consulté sur le DUERP et ses mises à jour. Consulter les représentants du personnel quant à l'évaluation des risques professionnels contribue effectivement à la qualité du dialogue social et à la pertinence du programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

du CSE. Par ailleurs, si l'élaboration du DUERP s'inscrit dans une démarche de consultation des instances de dialogue social de l'entreprise, il s'agit d'un document dont la responsabilité incombe au seul employeur, qui doit rester maître de son contenu. Quel est l'avis du

sur les questions de santé et de sécurité, tels qu'une commission paritaire dédiée à la santé et à la sécurité au travail, en particulier quand leur comité technique national et les autres instances existantes ne permettent pas de répondre totalement aux besoins.

Poumirol. Dans sa version actuelle, l'article 2 de la proposition de loi prévoit que le DUERP et ses versions successives sont tenus à la disposition des travailleurs et des anciens travailleurs.

monsieur le rapporteur,

l'entreprise. Dans sa version actuelle, l'alinéa 24 prévoit que le DUERP et ses versions successives sont conservés par l'employeur et tenus à la disposition des travailleurs - il faut entendre ce que cela signifie

En ce sens, une simple tenue à disposition du document ne suffit pas. Tout ancien travailleur qui en fait la demande doit se voir remettre un extrait du document unique. Tel est le sens de cet amendement.

Dans sa version actuelle, l'alinéa 24 de l'article 2 prévoit que le DUERP et ses versions successives sont conservés par l'employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs, ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier un intérêt à y avoir accès, et ce pour une durée qui ne peut être inférieure à 40 ans. Si la mention d'une durée minimale de conservation constitue une avancée, la durée retenue, de 40 ans, nous semble trop courte.

mais effectifs. Par ailleurs et principalement, dans l'esprit de l'ANI, l'accessibilité au DUERP vise à permettre aux salariés de constituer éventuellement- nous l'avons déjà signalé -un dossier de maladie professionnelle. Il est donc indispensable que la durée de conservation garantisse l'accès à ce document, y compris aux ayants droit des salariés décédés.

En outre, la durée de 40 ans correspond en moyenne à la durée d'une carrière professionnelle. À l'inverse, la durée de 50 ans nous paraît excessive. La commission émet

il en résulte une défaillance dans l'organisation générale de la prévention, parfois jugée optionnelle, et l'absence de mesures particulières adaptées aux situations vécues par les salariés.

En outre, nous ne mesurons pas tout à fait la portée de ces ajouts législatifs, en ce qui concerne notamment l'obligation de moyens et la responsabilité des employeurs. Bien évidemment, nous partageons l'objectif de renforcer la prévention dans ses différentes dimensions,

Mme Raymonde Poncet Monge. L'article 2 de la proposition de loi prévoit que, lors de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail, les échanges entre l'employeur et les représentants du personnel pourront porter sur la qualité des conditions de travail. Le syndicat CFE-CGC, signataire de l'ANI, nous a alertés sur le fait que cette rédaction, en faisant de ces échanges une simple possibilité, ne traduisait pas l'esprit de l'accord national interprofessionnel,

par les termes « qualité de vie et des conditions de travail ». Par cet amendement, le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires propose d'aller jusqu'au bout de cette mise en cohérence de l'article 2 de la proposition de loi

négocier en entreprise sur la qualité des conditions de travail lorsque cette négociation s'inscrit dans le cadre des dispositions supplétives du code du travail, c'est-à-dire lorsque les partenaires sociaux n'ont pas conclu d'accord de méthode sur le contenu et la périodicité de la négociation. Cet amendement, qui a déjà été rejeté par la commission, vise au contraire à rendre ce thème obligatoire. Nous considérons, quant à nous, qu'il n'est pas souhaitable de contraindre excessivement la négociation en entreprise, au-delà des thèmes déjà imposés par le code du travail. Avis défavorable.

du travail, qui est souvent un facteur de risques psychosociaux. Redonner aux salariés, premiers concernés, la possibilité d'intervenir et de s'exprimer sur cette organisation est indispensable pour lutter efficacement contre les risques psychosociaux et redonner sens et utilité aux missions exercées. Nous proposons donc, par cet amendement, d'ajouter l'organisation du travail aux items sur lesquels la négociation en entreprise doit porter. Quel

Les actions de maintien dans l'emploi ou en emploi ont pour objectif de permettre à des personnes dont le handicap ou les problèmes de santé restreignent l'aptitude professionnelle à rester en activité ou à reprendre leur activité dès consolidation, soit par un aménagement de leur emploi soit par un changement d'activité ou d'emploi. Les estimations font état d'une fourchette située entre un et deux millions de salariés menacés à court ou moyen terme par un risque de désinsertion professionnelle, soit 5 à 10 % des salariés. C'est énorme ! de la désinsertion professionnelle se pose celle de l'aptitude professionnelle : actuellement, les salariés les plus concernés sont globalement moins qualifiés et plus âgés que les autres, les métiers ouvriers et des secteurs sanitaires et sociaux Si le Gouvernement a repris la recommandation de la mission préconisant de mieux définir les ambitions d'une politique de prévention de la désinsertion professionnelle, nous ne comprenons pas pourquoi celle-ci n'a pas été retenue En effet, l'IGAS proposait en même temps d'adopter une vision globale orientée vers la sécurisation des parcours professionnels en renvoyant vers la négociation collective et les services de santé au travail. Tel est l'objet de notre amendement.

et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Ce thème inclut donc déjà la prévention de la désinsertion professionnelle. Cet amendement, de notre point de vue, est satisfait. J'en demande donc retrait. À défaut,

Cet article, inséré en commission par l'Assemblée nationale, vise à prendre en compte les situations de polyexpositions pour les travailleurs exposés à des risques chimiques. Lors de l'examen de ce texte par la commission des affaires sociales du Sénat, certaines modifications ont été adoptées de prévoir que la visite post-exposition ait lieu dans les meilleurs délais après la cessation de l'exposition, et non plus seulement avant le départ à la retraite. Or le suivi individuel renforcé permet déjà d'assurer un suivi médical périodique pour les salariés exposés à des risques. Le médecin délivre alors un avis d'aptitude ou d'inaptitude, et propose à l'employeur des mesures individuelles telles qu'une mutation ou une transformation de poste. Le temps consacré aux visites et aux examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est bien évidemment compris dans les heures de travail du salarié sans qu'aucune retenue de salaire ne puisse être opérée, ou est rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent pas avoir lieu pendant les heures de travail. Afin d'éviter que ces nouvelles dispositions ne fassent doublon avec les mesures déjà existantes et afin de garantir la lisibilité de la loi, cet amendement tend à supprimer les alinéas prévoyant ce suivi post-cessation d'exposition. Quel

couvre toute sa période d'exposition ; le suivi post-exposition vise, quant à lui, à surveiller l'état de santé du travailleur après la cessation de cette exposition. Le suivi post-exposition s'inscrit dans la continuité du suivi individuel renforcé : il n'intervient donc pas en doublon de celui-ci. Supprimer la possibilité pour le médecin du travail d'engager une surveillance de l'état de santé du travailleur après la cessation de l'exposition priverait le travailleur d'actions de prévention, notamment de dépistage, contre des pathologies pathologies différées. Du reste, ce suivi post-exposition s'inscrit dans la même logique que la surveillance post-professionnelle, introduite par le Sénat en 2018 sur l'initiative de notre collègue Alain Milon, qui intervient avant le départ à la retraite des travailleurs exposés à des risques dangereux pour la santé.

quelque peu surprise par cet amendement : le suivi post-exposition à des risques dangereux est une avancée tangible et concrète pour les salariés les plus exposés à des risques professionnels.

que les travailleurs et travailleuses ont effectuées dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques professionnels ainsi que les attestations, certificats et diplômes obtenus dans ce cadre. L'existence d'un tel document suscite des craintes chez les professionnels comme chez certains partenaires sociaux, qui s'interrogent sur ses finalités, au-delà de l'intérêt de la traçabilité des formations continues suivies par le salarié. En effet, si chaque entreprise a par définition connaissance des formations qu'elle organise, il est de la libre décision de chaque salarié de porter à la connaissance d'un de ses employeurs l'ensemble des formations suivies au cours de son parcours professionnel comme de consentir à la transmission des informations qui font l'objet de ce passeport. Mais le refus d'en permettre l'accès peut engendrer un risque de discrimination, à l'embauche notamment.

Ces risques sont à mettre en regard d'une utilité très limitée par rapport aux dispositifs existants : tout salarié, s'il le souhaite, peut d'ores et déjà mentionner des formations à son employeur et, le cas échéant, fournir ses certificats ou attestations. Nous proposons donc de supprimer cet article.

collective vers une responsabilité individuelle du travailleur, celui-ci étant censé se former pour s'adapter à des conditions de travail éventuellement néfastes pour sa santé. santé. On assiste ainsi à une inversion de la logique et de la démarche de prévention, celle-ci consistant à agir prioritairement sur les conditions de travail et l'organisation du travail.

Il s'agit de renommer le passeport de prévention « livret de formation santé sécurité » afin de lever toute ambiguïté quant à la responsabilité personnelle de l'employeur. En effet, l'intitulé « passeport de prévention » présente deux limites aux yeux des membres de ce collectif. Tout d'abord, il ne rend pas compte du contenu du document créé à l'article 3 de la proposition de loi : ce document comprend uniquement des attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail, que celles-ci aient été dispensées par l'employeur ou par un organisme de formation, que le salarié les ait ou non suivies de sa propre initiative. De ce fait, le terme « livret de formation santé sécurité » paraît plus approprié et largement suffisant. Ensuite- cela a été rappelé -, nous craignons que l'intitulé « passeport de prévention » ne participe d'une logique de transfert d'une partie de la responsabilité de l'employeur vers le salarié.

Prévention AT-MP alerte sur un risque d'instrumentalisation du passeport de prévention visant à faire porter une partie de la responsabilité sur le salarié alors même que, subordonné,

réel. De nouveaux dispositifs étant créés, il convient de réaffirmer explicitement la responsabilité personnelle de l'employeur quant à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. C'est lui, l'employeur, qui doit veiller à l'effectivité de l'application des règles de sécurité,

Ce collectif dénonce une déresponsabilisation des employeurs et une régression historique dans le champ de la prévention des risques professionnels, dont le fondement juridique serait profondément remis en cause. En effet, sous réserve qu'il réponde à un protocole, l'employeur sera quasiment déchargé de ses obligations à l'égard de la santé de ses salariés,

Deux jugements, en 2015 et en 2016, ont relativisé cette jurisprudence en transformant l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en obligation de moyens.

Pourtant, les obligations de formation et d'information ne correspondent qu'à une partie seulement de l'obligation qui incombe à l'employeur en matière de mesures de prévention. Ce livret de formation ne saurait suffire

l'alinéa 3, c'est-à-dire l'intégration du passeport de prévention au passeport d'orientation, de formation et de compétences. L'idée n'est pas de remettre en cause le principe général : c'est surtout une histoire de calendrier. Sur ce sujet, en effet, la négociation avec les partenaires sociaux n'est pas aboutie, ce qui occasionne pour eux de fortes difficultés.

précédemment à propos de l'amendement n° 99 : nous considérons que les formations, les attestations, les certificats et les diplômes listés dans le passeport de prévention n'exonèrent pas l'employeur de sa responsabilité quant à la préservation de la santé des travailleurs. En effet, les organisations syndicales et les associations d'accidentés du travail s'inquiètent très fortement et légitimement des conséquences de la création de ce passeport de prévention.

Pour autant, il est nécessaire de mettre en place et d'évaluer le dispositif innovant du passeport de prévention avant de procéder, le cas échéant, à son élargissement par voie réglementaire.

Ces amendements tendent à renommer le passeport de prévention « livret de formation santé sécurité ». Ils visent en outre à préciser que ce livret ne peut se substituer aux obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité vis-à-vis du travailleur.

en matière de santé et de sécurité au travail : il doit permettre d'identifier les compétences qui ont été acquises et celles qui restent à acquérir ou à renouveler pour assurer un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité du travailleur.

qu'ils auront suivies en matière de santé et de sécurité au travail. Ce sera un outil puissant de réinsertion professionnelle pour le demandeur d'emploi, qui pourra faire valoir les habilitations acquises, mais également de visibilité pour l'employeur, celui-ci connaîtra les obligations de formation déjà satisfaites, évitant ainsi un certain nombre de redondances dans les formations qu'il devra organiser pour le candidat si celui-ci est retenu. Ce dispositif est issu des auditions que nous avons menées, Pascale Gruny et moi-même.

Le rôle de conseil des services de santé au travail était déjà possible, tant auprès de l'employeur que des salariés, tout en devant rester centré sur ses missions propres, rappelées dans un avis du Conseil d'État, à savoir « d'éviter toute altération de la santé du travailleur du fait du travail ».

de baisse de la démographie de praticiens en médecine du travail, de temps hypercontraint et de manque structurel de moyens, le fait de faire peser sur les SST des missions relevant de la médecine générale ou de la santé publique

qui ont réformé ces services pour recentrer leurs missions sur la santé au travail autour d'une offre socle obligatoire. Pour que cette offre socle soit effective, dans le dans le contexte de pénurie que nous connaissons, il est essentiel de centrer l'action des SPSTI sur leurs trois missions de base, à savoir la prévention,

Les nouvelles façons de travailler, avec l'essor du télétravail, ont eu comme corollaire de déconnecter un certain nombre de salariés de leur réseau professionnel. Le travail émancipe, mais ne protège pas toujours les femmes. La généralisation du télétravail équivaudrait, dans l'état actuel de nos sociétés, à une aggravation des inégalités entre hommes et femmes. Les filets de sécurité associés au monde professionnel dans les entreprises les avantages de prémunir, voire de réduire, des actes éventuels de violence commis à l'encontre des femmes. Le rôle du médecin du travail s'avère donc structurant dans ce type de situations de confinements à répétition. Cet amendement vise à faire du personnel de santé au travail un nouvel acteur dans la lutte contre les violences conjugales et sexuelles. Ces professionnels sont des rouages essentiels dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

à savoir la prévention des risques professionnels, le suivi médical et la prévention de la désinsertion professionnelle et, d'autre part, les missions complémentaires du SPST, qui tiennent à sa contribution à l'atteinte d'objectifs de santé publique qui doivent permettre de maintenir le travailleur dans un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette clarification entre des missions principales de santé au travail et des missions complémentaires de santé publique a été demandée par le Conseil d'État. Il n'y a pas de risque que le SPST néglige ses missions essentielles au titre de l'offre socle, puisque la certification et l'agrément doivent justement prévenir de telles dérives. Estimant que la rédaction issue des travaux de la commission répond aux inquiétudes

bien qu'il ait pour objet la prévention des violences conjugales ou sexuelles, il échappe aux « fourches » de l'irrecevabilité au titre de l'article 45 de la Constitution en empruntant la voie d'entrée de la contribution SPST à la promotion de la santé dans le cadre d'objectifs de santé publique, possibilité que prévoit effectivement l'article 4 de la proposition de loi dans sa version initiale. Toutefois, l'amendement reste problématique pour des raisons principalement de deux ordres. D'une part, son adoption allongerait l'énumération figurant au dernier alinéa de l'article 4 des actions de sensibilisation que le SPST peut mettre en oeuvre, énumération qui pourrait être poussée à l'infini. Dans un souci d'intelligibilité de la loi, il est préférable de ne pas complexifier outre mesure cette énumération qui a déjà été considérablement alourdie par l'Assemblée nationale. D'autre part, l'amendement vise à mettre l'accent non seulement sur la sensibilisation aux violences sexuelles qui prennent leur origine sur le lieu de travail, mais aussi sur la sensibilisation aux violences conjugales. Cette disposition découle de la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail des violences domestiques sur les conditions de travail. Nous ne nions bien entendu pas cet impact, mais il convient d'être prudent : il faut garder à l'esprit que le sujet des violences conjugales met potentiellement en jeu le partage très délicat d'informations personnelles et familiales, pour lequel le le cadre de la promotion de la santé sur le lieu de travail par le SPST ne paraît pas pertinent. Les salariés peuvent déjà solliciter aujourd'hui l'assistant social ou le psychologue du service de santé au travail pour aborder des problèmes qui dépassent la sphère professionnelle : il est donc préférable de privilégier ce cadre plus protecteur de la confidentialité des informations personnelles du salarié concerné. Pour l'ensemble de ces raisons, je demande le retrait de cet amendement.

que les anciens CHSCT permettaient d'analyser, d'où le vide laissé par leur suppression. Si nous sommes d'accord sur le fait que cette proposition de loi ne doit pas aboutir à une déresponsabilisation des employeurs,

dans la démarche d'évaluation des risques. Ces missions sont l'objet d'enjeux très forts pour l'employeur. Actuellement, le droit protège le médecin du travail, et lui seul, lui seul, du licenciement lors du renouvellement d'un CDD ou d'un transfert vers une autre entreprise. De même, la prérogative du médecin d'imposer son signalement de risque et ses préconisations à l'employeur, qui doit y répondre, le légitime, seul, dans ses missions d'évaluation des risques et de prévention.

de la bonne exécution de l'évaluation des risques. L'aide du service de prévention et de santé au travail ne remet pas en cause la responsabilité entière de l'employeur dans l'évaluation des risques, ainsi que dans la définition et la mise en oeuvre des mesures de prévention. Alors que le Gouvernement souhaite élargir les missions des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail à l'accompagnement dans l'évaluation des risques professionnels et à la promotion de la santé sur le lieu de travail, les professionnels demandent une meilleure protection. Actuellement, le droit protège les médecins du travail dans leurs missions d'évaluation des risques et de prévention. Or, on l'a dit, mais il convient selon moi de le répéter, la réduction du nombre de médecins du travail et l'extension des missions de prévention à l'ensemble des équipes pluridisciplinaires des services de prévention nécessitent de renforcer leur protection et leurs prérogatives.

les amendements visent à étendre à tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire du SPST le statut de salarié protégé, qui est aujourd'hui réservé au médecin du travail, médecin de l'aptitude. La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficie le médecin du travail en tant que salarié protégé est liée aux fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs. Les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire exerçant leurs missions sous l'autorité du médecin, il n'y a pas lieu de leur étendre le statut de salarié protégé.

cette mission relève de la santé publique. Alors que les services de prévention et de santé au travail font face à une pénurie de moyens et de médecins du travail,

inégalité de traitement entre les salariés. En effet, les campagnes de vaccination et de dépistage pourraient être à géométrie variable, selon la taille de l'entreprise ou le lieu de travail. En outre, l'employeur pourrait avoir connaissance d'informations sensibles sur l'état de santé du salarié, par exemple des résultats de test PCR, une pratique déjà en cours dans le contexte de pandémie de covid-19. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression

Bien sûr, la santé au travail participe de la santé publique, mais ses objectifs ne doivent pas être dilués dans ceux de la santé publique. C'est pourquoi il convient de circonscrire

ce qui, de notre point de vue, va dans le bon sens. La mise en oeuvre de campagnes de vaccination et de dépistage y participe, comme l'a rappelé M. le secrétaire d'État. La pandémie a démontré que le risque infectieux se posait dans tous les milieux de vie, tout particulièrement sur le lieu de travail. En outre, l'origine multifactorielle de certaines pathologies, notamment cancéreuses, liées à des facteurs professionnels et environnementaux, plaide pour une sensibilisation renforcée des travailleurs au bénéfice des dépistages.

s'entendent, bien entendu, comme des missions complémentaires des SPST, dont la vocation principale, comme l'a rappelé la commission des affaires sociales, est de prévenir l'altération de l'état de santé du fait du travail. En outre, nous avons précisé à l'article 8 que l'offre socle obligatoire des SPST comprenait trois champs : le suivi individuel du travailleur, la prévention des risques professionnels, la prévention de la désinsertion professionnelle. La promotion

l'énumération des actions de sensibilisation possibles, laquelle pourrait être poussée à l'infini. Dans un souci d'intelligibilité de la loi, il est préférable de ne pas complexifier outre mesure

le rôle des SPST dans la sensibilisation aux troubles auditifs. La proposition de loi prévoit déjà que les SPST pourront mettre en oeuvre des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap, ce qui comprend

le sujet des violences conjugales met potentiellement en jeu le partage très délicat d'informations personnelles et familiales, pour lequel le cadre de la promotion de la santé sur le lieu de travail par le SPST ne paraît pas pertinent. Les salariés peuvent déjà solliciter

puisqu'il est fait référence au personnel de santé au travail, sans qu'il soit précisé s'il s'agit du personnel recruté par le service de prévention et de santé au travail ou d'intervenants extérieurs auxquels le SPST pourrait avoir recours.

Dans le prolongement de l'obligation de prévention qui incombe aux employeurs, cet amendement vise à permettre le suivi post-professionnel par les services de prévention et de santé au travail des salariés licenciés pour une inaptitude d'origine professionnelle. Alors qu'un projet de décret modifiant les modalités du suivi post-professionnel des salariés, afin d'en simplifier l'accès, a été soumis à la mi-juin 2021 au Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT), il semble indispensable que les salariés à la retraite, au chômage ou inactifs puissent bénéficier d'une surveillance médicale, dès lors qu'ils ont été exposés à des produits à effets différés sur la santé. Jusqu'à présent, un salarié devait présenter une attestation d'exposition cosignée par l'employeur et le médecin du travail pour bénéficier d'un suivi post-professionnel.

Quel est l'avis de la commission ? Le suivi de l'état de santé des demandeurs d'emploi est un véritable enjeu de santé publique, que l'on sous-estime et qui reste l'angle mort de la médecine de prévention. Certaines études montrent qu'ils sont proportionnellement plus touchés par les maladies chroniques, addictions, voire les suicides. Pour autant, le suivi post-professionnel des personnes licenciées pour inaptitude ne peut pas être confié aux SPST dont le public recouvre, par définition, les salariés employés par les entreprises qui leur sont affiliées. C'est à ce titre que les ressources des SPST reposent sur les cotisations versées par les employeurs, lesquelles sont calculées en fonction de leurs effectifs salariés. Par ailleurs, les SPST se sont vu reconnaître une mission dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, pour mieux anticiper l'impact sur la carrière des risques d'inaptitude. Les actions menées à ce titre doivent permettre de favoriser le maintien en emploi des personnes concernées. Par conséquent, la

le professeur Paul Frimat, spécialiste de médecine du travail, a rendu, en 2018, un rapport relatif à la prévention et à la prise en compte de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux.

Pris de manière globale, ce changement de méthode est une réduction des coûts pour la sécurité sociale et un gain d'expertise pour les travailleurs, y compris les retraités. Ce suivi par la médecine du travail permettrait également de circonscrire l'anxiété et la difficulté de faire reconnaître le lien entre exposition et complications. Il s'agit d'un progrès pour l'ensemble des travailleurs, qui, par effet rebond, renforce également la responsabilité des employeurs, lesquels sont chargés de limiter les expositions aux produits considérés

par l'article L. 4624-2-1 du code du travail, de procéder à un examen médical de chaque travailleur bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé au titre de l'exposition à des risques particuliers avant le départ à la retraite. S'il constate une exposition à certains risques dangereux, notamment chimiques, le médecin du travail a la faculté de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant du travailleur. Cet amendement étant satisfait par le droit en vigueur, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle

La constitution par la médecine du travail d'un dossier médical en santé au travail est obligatoire pour chaque salarié suivi. La commission des affaires sociales a, en outre, rappelé à l'article 12 que devront être consignées dans le dossier médical en santé au travail (DMST) toutes les données d'exposition à des risques professionnels de nature à affecter l'état de santé du travailleur.

Alors que, selon les derniers résultats de CoviPrev, 19 % des Français souffrent d'un état dépressif et 21 % d'un état anxieux, il paraît essentiel que les services de prévention et de santé au travail se saisissent des sujets de santé mentale. En effet, la notion de burn-out a fait son apparition dans notre langage courant depuis quelques années. Ce syndrome d'épuisement professionnel est un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique. La santé mentale, qui est essentielle à la santé au travail,

relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) et au règlement européen relatif à la surveillance du marché. Cet amendement vise à préciser et à compléter ces dispositions sur le volet des pouvoirs et des habilitations des administrations compétentes, l'objectif étant de remédier à des non-conformités de conception et d'éviter ainsi la survenance ou la reproduction des accidents, grâce à l'action de contrôle de l'administration.

Poncet Monge, pour présenter l'amendement n° 56. L'article 8 crée une offre socle et une offre complémentaire pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), ainsi qu'une procédure de certification par des prestataires privés pour contrôler le service rendu. Tout d'abord, le principe même d'une offre complémentaire est problématique. Introduire une distinction entre une offre socle et une offre complémentaire nous paraît dangereux et inapproprié, compte tenu de l'objet même des services de santé au travail : éviter éviter toute altération de la santé des salariés en lien avec leur travail. La santé et la sécurité des travailleurs ne sauraient comporter des composantes optionnelles. De plus, cela entraînera une rupture d'égalité entre les travailleurs, selon que leur employeur contracte ou non une offre complémentaire. Comme toute création d'une offre « à plusieurs vitesses »- faut-il rappeler les précédents ? -, l'expérience nous enseigne que la dynamique conduit à bloquer l'offre socle, voire à la réduire, au profit d'un étoffement de l'offre complémentaire, productrice de recettes elles-mêmes complémentaires pour les services de santé au travail. Par ailleurs, comment cette offre complémentaire trouverait-elle des ressources humaines sans empiéter sur l'offre socle, alors que nous constatons l'espacement continu des visites, notamment pour des raisons de pénurie de professionnels comme d'objectif de baisse des coûts pour les employeurs ? Enfin, le contrôle par des prestataires privés de la qualité du service rendu, y compris de son efficacité, nous paraît présenter un risque. En effet, la définition du cadre et des objectifs

dits , qu'en sera-t-il pour les autres ? Quels services seront considérés comme facultatifs ? Ce texte peut ainsi déboucher sur un système de santé au travail à deux vitesses. L'instauration d'une dichotomie entre offre socle de services et offre de services complémentaires peut conduire à des inégalités de traitement entre les salariés

toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 8. l'avis de la commission ? La définition d'un ensemble socle de services et la mise en place d'une procédure de certification font partie des mesures structurantes prévues par l'ANI du 9 décembre 2020 et reprises par la proposition de loi, pour améliorer la qualité des services rendus par les services de prévention et de santé au travail interentreprises. La commission a adopté cet article en lui apportant des améliorations, notamment des garanties sur le contenu de l'offre socle et une capacité d'initiative des partenaires sociaux sur le cahier des charges de la certification. Par conséquent, elle ne peut

parole est à M. Joël Guerriau. La proposition de loi confère de nouvelles prérogatives au service de prévention et de santé au travail (SPST) : aide à l'évaluation des risques, mise en place d'une offre de services complémentaire pour les salariés, mise en place d'une offre spécifique dédiée aux travailleurs indépendants.

en prévention des risques professionnels (IPRP) externes pour des missions spécifiques. Nous reconnaissons, bien sûr, le rôle important de ces intervenants, mais le fait de l'inscrire dans la loi n'améliorera pas le droit existant.

De plus, il ne paraît pas souhaitable que les comités régionaux de prévention et de santé au travail aient à se prononcer à ce sujet. Bien que leur rôle prévoie l'élaboration des référentiels de certification, celui-ci ne comprend pas qu'ils se prononcent sur une procédure administrative individuelle.

la procédure d'agrément administratif des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI). La commission a proposé, en cohérence avec la réforme de la gouvernance territoriale de la santé au travail, que le comité régional de prévention et de santé au travail (CRPST), institué par la proposition de loi au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail (Croct), formule formule un avis sur cet agrément pour les SPSTI relevant de son ressort territorial. Le CRPST est notamment composé de représentants des organisations syndicales et patronales représentatives.

qui travaillent dans l'entreprise. Actuellement, les employeurs ont l'obligation d'avoir recours à un service de santé au travail autonome ou intégré, dont les missions sont définies, contrairement à ce que prévoient l'offre socle Cela pose un problème d'égalité entre les salariés, qui bénéficieront d'une protection différente selon l'entreprise dans laquelle ils seront embauchés et selon le degré de protection que cette entreprise pourra offrir. En renvoyant la certification à des organismes indépendants privés non identifiés, vous privatisez l'action publique en matière de santé au travail.

Cet article porte atteinte à la philosophie même du rôle des médecins du travail, qui ne veulent pas mener une intervention si l'entreprise n'a pas souscrit à l'offre.

Lors de vos travaux en commission, vous avez modifié les attributions du comité national de prévention et de santé au travail en lui confiant un rôle de proposition, et non plus d'avis, sur les référentiels et les principes qui guident l'élaboration du cahier des charges de certification.

La commission a prévu de laisser aux partenaires sociaux, par l'intermédiaire du CNPST, l'initiative de la détermination du cahier des charges de la certification introduite par l'article 8.

devant le constat partagé d'une forte hétérogénéité des services rendus par les SCCI, d'améliorer leur qualité et leur effectivité. C'est véritablement ce qui a animé la On ne peut en effet se satisfaire de la procédure existante d'agrément administratif, dont la portée est en pratique très limitée. La procédure sera encadrée par des référentiels fixés par l'État, sur lesquels les partenaires sociaux auront leur mot à dire au travers du CNPST.

dans la détermination du cahier des charges de la certification, réduisant ce rôle à un simple avis pour le CNPST. Le sous-amendement de la commission revient sur ce point. D'autre part, le décret serait publié au plus tard le 30 juin 2022.

sa dissolution. Des services de santé continuent donc de fonctionner en l'absence d'agrément. Par ailleurs, il arrive que certaines Direccte ne soient pas en mesure de refuser un agrément, du fait du monopole territorial du service examiné. Il paraît donc nécessaire de prévoir la possibilité de prendre d'autres mesures afin de contraindre les services à mettre un terme à leurs dysfonctionnements, compte tenu des conséquences que ceux-ci ont sur les salariés suivis. Par cet amendement, nous proposons que l'autorité administrative puisse sanctionner financièrement ces services et, beaucoup plus largement, que toute autre sanction puisse être prise pour mettre fin aux dysfonctionnements. Ainsi, l'autorité administrative pourrait ordonner le regroupement d'un service non efficient avec un service voisin, voire révoquer le président du service. Cette proposition va dans le sens voulu par les partenaires sociaux signataires de l'ANI, qui se sont prononcés pour des sanctions graduées. Quel

un système d'administration provisoire des services de prévention et de santé au travail dans les situations où des défaillances graves en termes d'organisation sont constatées n'en fait absolument pas partie.

Afin de doter l'administration d'un moyen d'action plus efficace et constructif que le retrait d'agrément en cas de difficulté grave d'organisation et de fonctionnement, la commission a proposé l'introduction d'un régime d'administration provisoire qui doit permettre, sans interrompre le service, de lui donner les moyens de se réorganiser. Ce dispositif est inspiré du régime applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il s'agit bien entendu d'un instrument qui serait utilisé par l'administration

juridiquement possible de mettre sous administration provisoire une structure associative de droit privé qui relève de la loi de 1901. Je ne

et sociale. Avec les restrictions d'aptitude, elles concernent tous types de public, dont un grand nombre ne sont pas reconnus comme travailleurs handicapés. Cela va dans le sens de l'inclusion. La prise en charge de ce type de dossier est chronophage : ces situations demandent un suivi important qui ne peut être réalisé par le médecin du travail, par manque de temps, de connaissance des acteurs et des dispositifs qui évoluent constamment. En fonction des besoins, les chargés de mission de la prévention de la désinsertion professionnelle et du maintien en emploi pourront prendre ces dossiers en charge et, à ce titre, faire partie de l'équipe médicale. Dans ce cadre, ils devraient être pris en compte dans l'offre socle, tout comme les infirmiers ou les assistantes sociales. La prise en compte de ces situations et leur traitement par les chargés de mission permettent de limiter les licenciements grâce à la mise en oeuvre d'aménagements, d'organisations spécifiques ou d'orientations précoces,

Sur le territoire, plusieurs services de prévention et de santé au travail ont fait la démonstration de l'efficacité de la présence de chargés de mission pour maintenir en interne des personnes en activité. Cela se vérifie notamment pour les services ayant une forte pénurie de médecins du travail.

Toutefois, rien n'empêche aujourd'hui les services de prévention et de santé au travail de créer des équipes de chargés de mission, qui sont d'ailleurs efficaces. Inscrire cette possibilité dans la loi ne permet pas d'améliorer le droit existant.

M. Joël Guerriau. L'accord national interprofessionnel sur la santé au travail, signé le 9 décembre 2020 par les partenaires sociaux, considère que la branche professionnelle est un cadre privilégié pour formaliser pour formaliser les grandes priorités dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Cet accord précise, par ailleurs, que les services de santé au travail de branche, qui participent activement à la prévention des risques professionnels dans les secteurs concernés, doivent conserver leurs spécificités. Dans ces conditions, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services de branche intègrent les priorités par branche professionnelle. En complément, dans un secteur spécifique comme le BTP, doté de différentes structures « santé prévention », il est nécessaire pour la bonne articulation entre les acteurs que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) soit également conclu avec l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), dont l'existence, l'organisation et le déploiement

quadripartite incluant la signature de l'organisme professionnel de prévention du BTP, l'OPPBTP. Si l'OPPBTP peut légitimement avoir un droit de regard sur le cadre de l'action des services actifs dans le secteur du bâtiment, le dispositif proposé est source de complexification. De fait, cette pratique, prévue par une convention en

L'article 11 permet aux professionnels de santé des services de prévention et de santé au travail d'accéder au dossier médical partagé

l'intégrité des données personnelles de santé des salariés, dont le consentement ne saurait être totalement libre dans le cadre de la relation de subordination qu'est la relation de travail.

Si la médecine du travail doit avoir les moyens de juger des risques d'altération de la santé du salarié en lien avec son travail, notamment un suivi régulier du salarié et de ses conditions concrètes de travail, l'accès à l'ensemble du dossier médical serait disproportionné

D'une part, cette disposition entretient une confusion entre santé publique et santé au travail. D'autre part, cette mesure permettrait à la médecine du travail d'avoir accès aux données de santé sensibles contenues dans le dossier médical partagé des salariés, ce qui pose la question de la confidentialité de ces données. Si la santé publique doit s'intéresser à la santé au travail,

nourrissons des inquiétudes notamment pour les informations confidentielles des personnes en affection longue durée. Je pense particulièrement à la séropositivité et à la transition des personnes transgenres ; nous craignons que ces personnes ne fassent ensuite l'objet de discriminations.

En effet, permettre au médecin du travail d'accéder à ces données, même avec l'accord du patient, risque d'être préjudiciable au salarié, en particulier lors des visites d'embauche et de reprise du travail,

Le médecin du travail est aussi conduit à se désintéresser des maladies professionnelles, comme ce fut le cas pour l'amiante, et à focaliser son attention sur les aptitudes propres du salarié à remplir les missions qui lui sont dévolues, Nous insistons donc sur la nécessité que le médecin du travail dispose simplement d'un accès spécifique et cloisonné au DMP, lui permettant de consigner les comptes rendus de visite, l'exposition à d'éventuels risques, les aménagements des situations de travail et les contre-indications médicales, mais rien de plus et surtout sans

du travailleur, avec, bien entendu, le consentement de ce dernier et dans le respect de la plus stricte confidentialité des données. Les modifications apportées par la commission des affaires sociales visent précisément à renforcer cet encadrement, afin de préserver la confiance et la relation

de suppression de l'article 11, qui permet au médecin du travail d'accéder au dossier médical partagé après accord du salarié. À défaut de supprimer l'accès à ce dossier, il convient de garantir au mieux l'expression du libre consentement du salarié au partage de ses données personnelles

C'est pourquoi la commission des affaires sociales a modifié l'article 11 pour prévoir que ce consentement ne pourra pas être donné oralement, mais devra emprunter une voie dématérialisée préservant le libre choix du travailleur.

est renvoyée à la prochaine séance. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative